Madame la présidente,

je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents. J'invite par ailleurs chacune et chacun d'entre vous à veiller au respect des gestes barrières.

Le 25 mars 2020, à Mulhouse, le Président de la République avait annoncé un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières dans les hôpitaux.

Il a ainsi créé des différences de traitement entre les professionnels du soin. Les nombreux exclus du Ségur ont vécu ces annonces comme un manque de considération à leur égard. Ces professionnels du soin sont nombreux et divers : ils sont infirmiers, éducateurs, assistants sociaux, aides-soignants, agents administratifs, psychologues, puéricultrices, intervenants éducatifs, sages-femmes, ou encore ambulanciers. Ils travaillent dans des structures aux statuts variés : associations, fondations, entreprises privées, collectivités territoriales. Prendre soin des Français, c'est aussi prendre soin de publics divers : des personnes fragiles, âgées, handicapées, des enfants en danger. Au gré des sollicitations plus ou moins fortes de chacune de ces catégories, le Gouvernement a ajouté de nouveaux bénéficiaires au Ségur en procédant par touches successives.

Pour Marie-Reine Tillon, présidente de l'Union nationale de l'aide à domicile, il est hors de question de revoir à la baisse le montant négocié pour revaloriser la convention collective de la branche. Il faut donc trouver les ressources correspondantes.

Ce manque de personnel aboutit à des plans d'aide réduits et à des refus de prise en charge de personnes âgées, notamment à domicile. Nous saluons néanmoins les annonces faites en cette fin d'année, qui visent à étendre les revalorisations salariales accordées lors du Ségur de la santé aux professionnels du secteur du handicap, qui concernera 20 000 soignants. Alors qu'il faudra plus de 90 000 infirmiers et plus de 200 000 aides-soignants dans les prochaines années pour accompagner les 5 millions de Français de plus de 85 ans, comment faire face à

Madame la ministre, pouvez-vous nous en dire plus sur la tenue de cette conférence et les orientations que proposera le Gouvernement, sur les compensations financières versées aux employeurs mis en difficulté, ainsi que sur l'extension à tous les personnels du soin des revalorisations salariales du Ségur de la santé ? La

pertinent que jamais de faire le point sur les actions menées par le Gouvernement pour les soutenir dans le cadre du Ségur de la santé. Je le souligne d'entrée de jeu : après plus de dix ans de sous-investissement dans les ressources humaines et les structures de l'hôpital public, le Ségur de la santé est de loin le plus important plan de soutien à notre système de soins jamais proposé par une majorité présidentielle. Cette ambition, c'est d'abord celle du Président de la République qui a pris à Mulhouse, le 25 mars 2020, l'engagement devant la Nation entière d'un plan massif d'investissement. Le Gouvernement a concrétisé cette promesse

revaloriser les métiers et les carrières de ceux qui soignent ; définir une nouvelle politique d'investissement massive ; simplifier le quotidien et l'organisation des équipes de santé ; enfin, fédérer les acteurs de santé dans les territoires au service des usagers. Commençons par les carrières des personnels soignants, des médecins et des professionnels de santé. La première urgence à laquelle nous nous sommes attelés était de reconnaître et de revaloriser leurs compétences. À travers les accords du Ségur signés par le Premier ministre le 13 juillet 2020,

d'une revalorisation socle de 183 euros par mois. Je dis bien « au moins », puisque, depuis octobre 2021, nous avons également revalorisé les grilles des personnels soignants, médico-techniques et du secteur de la rééducation. Aides-soignants, infirmiers spécialisés ou non, cadres de santé, kinésithérapeutes, manipulateurs radio, ergothérapeutes, psychomotriciens, et j'en passe : tous sont concernés. Parlons concrètement : le Ségur de la santé représente ainsi pour un infirmier de la fonction publique une revalorisation de 290 euros net en début de carrière, 335 euros après cinq ans de carrière, et 530 euros en fin de carrière. Les personnels médicaux ne sont pas en reste : nous avons fusionné les quatre

Concernant l'avenir de notre système de santé, nous avons revalorisé les indemnités de stage des étudiants en santé et des internes pour accompagner les vocations.

Toutes les professions ne sont pas concernées de la même manière par ce phénomène ni au même moment. C'est donc sur le fondement avéré de la perte d'attractivité des métiers que nous avons étendu à plusieurs reprises les revalorisations prévues, au-delà de l'ambition initiale, notamment à des personnels non médicaux. Le Premier ministre a confié dès l'automne 2020 à Michel Laforcade la mission de mener une réflexion et d'engager des négociations relatives à l'extension des revalorisations du Ségur aux professionnels paramédicaux des secteurs proches des deux protocoles ont été signés avec les organisations syndicales. Depuis le 1 octobre 2021, l'intégralité des personnels non médicaux des structures sanitaires et médico-sociales financées par l'assurance maladie bénéficie des 183 euros net Depuis le 1 janvier, ils ont été rejoints par les personnels des structures médico-sociales publiques et privées non lucratives qui interviennent dans le secteur du handicap ou des soins à domicile. Je le répète : nous avons cherché à donner l'ampleur la plus large possible à l'ambition initiale du Ségur de la santé.

des nombreuses et belles associations qui oeuvrent dans le champ des solidarités et de la santé. Ces deux chantiers sont distincts du Ségur de la santé et méritent d'être menés dans un cadre

La tenue de cette conférence a été retardée par le contexte sanitaire, mais elle aura lieu dans les prochaines semaines. Sa préparation a été confiée à deux experts, MM. Jean-Philippe Vinquant sociales (IGAS). Notre objectif est d'apporter des améliorations concrètes aux professionnels du secteur social et médico-social, tout en assurant une révision en profondeur des conditions d'exercice de leurs métiers et du déroulement de leurs carrières. Pour en revenir au Ségur de la santé, il représente des efforts considérables pour rendre les carrières des soignants plus attractives et témoigner de la reconnaissance de la Nation à leur égard, efforts qui ont culminé à près de 10 milliards d'euros de dépenses depuis la signature des accords en juillet 2020.

pour répondre aux ambitions que nous nous sommes fixées. Pour transformer notre système de santé dans les territoires, le Ségur prévoit 9 milliards d'euros d'aides visant à favoriser la réalisation de projets structurants pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, la construction de nouveaux bâtiments ou encore la rénovation de chambres d'hospitalisation pour améliorer le confort des patients. Enfin, le Ségur c'est aussi 2 milliards d'euros pour le numérique en santé. le Premier ministre, le ministre des solidarités et de la santé et moi-même avons lancé la stratégie nationale d'investissements en santé à Cosne-Cours-sur-Loire, avec le parti pris déterminé d'une déconcentration des enveloppes et d'une forte dimension territoriale, pour être au plus près des besoins en santé de nos bassins de vie. caractérisée par un changement de méthode et de vitesse sans précédent par rapport à ce qui se faisait auparavant. Il a ainsi été demandé aux ARS de mener en un temps record des concertations territoriales avec l'ensemble des acteurs de santé et des élus impliqués, pour définir les besoins selon une logique non pas d'établissements, mais de territoires de santé.

au profond malaise du monde de la santé : il ne répond ni au manque d'attractivité de ces professions ni à la dégradation de leurs conditions de travail. Quant aux investissements, qui consistent essentiellement en la reprise d'une partie de la dette hospitalière,

des organisations et des environnements de travail prévoit notamment l'instauration d'une prime d'engagement collectif de 100 euros net par mois pour promouvoir la participation des agents aux projets hospitaliers. Le Gouvernement a souhaité accompagner les établissements dans le recrutement de 15 000 personnels soignants, dans la rénovation des organisations de travail en incitant au dialogue social dans chaque établissement.

Dans ce contexte, vous avez pris des mesures très attendues par les acteurs de terrain, notamment la revalorisation des salaires des soignants et un investissement massif dans les hôpitaux, qui font l'objet de notre débat d'aujourd'hui.

pouvez-vous lever les inquiétudes qui minent les acteurs de cet établissement, les élus locaux et la population, et les assurer de la mobilisation de crédits en faveur de cet hôpital, lequel assure des missions de service public essentielles ?

une délégation, unique en son genre, d'un collectif rassemblant des employeurs et des syndicats de l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Ceux-ci s'étaient mobilisés en nombre dans tout le département du Finistère pour demander une revalorisation salariale de l'ensemble des professionnels du secteur médico-social

crée d'importantes iniquités au sein d'un même établissement, voire d'une même équipe, puisque les professionnels ne perçoivent pas tous le même traitement, malgré des fonctions et des qualifications analogues.

Au-delà du Ségur, c'est la faiblesse structurelle des salaires, la dégradation des conditions de travail et le manque de considération pour le secteur social et médico-social qui sont aujourd'hui en cause.

telle violence n'a pas sa place en démocratie, encore moins dans l'enceinte d'un hôpital. Permettez-moi de leur exprimer à nouveau mon amitié et de leur apporter tout mon soutien. Madame la ministre, sur les 14,5 milliards d'euros d'investissement prévus dans le cadre du Ségur de la santé pour les établissements de santé, plus de 1 milliard d'euros sera consacré aux outre-mer. Cette somme permettra d'améliorer la trésorerie des établissements, de les désendetter, au moins partiellement, et les aidera à assurer leurs investissements courants.

L'isolement géographique des outre-mer justifie, selon les conclusions du rapport de nos collègues Jean-Michel Arnaud et Roger Karoutchi, « un dimensionnement de l'offre de soins au moins équivalent à celui de l'Hexagone », notamment en ce qui concerne les capacités en soins critiques. La refonte du coefficient géographique et des modes de financement des hôpitaux ultramarins est la clef de cette autonomie ; elle permettra de réduire le nombre d'évacuations de patients vers l'Hexagone et les frais exorbitants que celles-ci emportent, mais également de constituer des pôles d'excellence.

Monsieur le sénateur Théophile, permettez-moi de vous remercier pour le soutien que vous apportez au directeur général du CHU de Guadeloupe, Gérard Cotellon, et à ses équipes. Les violences dont ils ont été la cible sont inacceptables, surtout dans le climat actuel ; nous devons afficher un front uni pour condamner ces actes commis à l'encontre de ceux qui assurent le fonctionnement des hôpitaux au service de la population. Comme vous, je les condamne avec la plus grande fermeté. Pour en revenir à votre question, l'agenda du Gouvernement n'a pas permis d'ouvrir une fenêtre propice à une discussion de type Ségur, pour

liberté, notamment, là où les dispositions métropolitaines ne paraissent pas adaptées. S'agissant du coefficient géographique, nous avons fait le choix de l'objectivité. Nous avons confié à la Drees la mission d'élaborer une méthode statistique robuste

Certes, les annonces gouvernementales constituent une réponse nécessaire et appréciée, mais elles demeurent insuffisantes. En se limitant aux soignants et aux personnels paramédicaux, elles excluent des professionnels pourtant indispensables à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, tels que les éducateurs spécialisés, les personnels administratifs, les agents de sécurité. Comme l'a indiqué M. le Premier ministre, « l'accompagnement des personnes en situation de handicap ne se résume pas aux soins De plus, cette situation sape les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap : ruptures d'accompagnement dues aux arrêts de service, problèmes de sécurité, restriction des activités essentielles à leur vie quotidienne, obligeant parfois les familles à

Monsieur le sénateur Franck Menonville, votre question porte sur l'action du Gouvernement dans le champ du handicap.

(CME) ont adopté une motion demandant l'application de cette nouvelle grille à tous. Ce dossier est à ce jour bloqué au niveau de votre ministère, alors que les représentants du secteur vous ont fait parvenir des propositions claires et efficaces pour fidéliser les praticiens hospitaliers.

000 praticiens bénéficient de ces primes managériales depuis novembre 2021 ; cela représente un engagement de plus de 80 millions d'euros. Au-delà du Ségur de la santé, le Gouvernement a pris des engagements en juillet dernier pour améliorer l'attractivité des carrières des personnels hospitalo-universitaires amélioration des rémunérations, mais aussi de la gestion des parcours professionnels, ou encore respect de l'égalité femmes-hommes dans l'accès à ces carrières. Au total, l'engagement du Gouvernement pour attirer et fidéliser des personnels non médicaux à l'hôpital représente un effort de près de 500 millions d'euros

mental et social. À ce cloisonnement s'ajoute un problème de périmètre, car ces revalorisations excluent de fait une grande partie du secteur social, par exemple le champ de la protection de l'enfance dont nous avons récemment débattu.

pour renforcer les dispositifs auprès des plus vulnérables durant les confinements successifs, assurer la continuité des actions de protection de l'enfance et faire face aux conséquences toujours en cours de la crise sanitaire et sociale. À l'heure où une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social est annoncée- elle est finalement reportée -, et où une mission est confiée à l'IGAS pour faire converger les conventions collectives du secteur, la ministre : le Gouvernement compte-t-il remédier avant la fin de son mandat, soit plus d'un an et demi après le début du Ségur, aux inégalités de traitement entre les professionnels de la santé, au sens de l'OMS, ainsi qu'aux dysfonctionnements induits par les distorsions d'attractivité

échanges révèlent des disparités de rémunérations qui aggravent les tensions au sein des équipes et suscitent un sentiment d'injustice, d'incompréhension et de colère.

dialogue entre les organismes financeurs de ces structures, l'État, les ARS, les départements et, plus largement, les collectivités et les associations ? Par ailleurs, la même disparité salariale existe entre les personnels des structures associatives et publiques. Quelles dispositions nationales d'harmonisation comptez-vous prendre pour éviter la fuite des travailleurs d'un secteur vers l'autre ? Enfin, les départements souhaitent disposer des modalités concrètes et d'un calendrier précis

dernier avait pour objectif d'améliorer et de revaloriser la carrière des personnels soignants de notre pays, mais il n'a apporté qu'une réponse partielle, seulement financière et en définitive insuffisante aux problématiques beaucoup plus globales que pose notre système de santé. la sécurité des patients est quotidiennement menacée. On assiste à de nombreux départs de soignants, écoeurés par leurs conditions de travail. Or c'est avant tout le manque de lits, de moyens et de personnel qui est pointé du doigt. à l'hôpital, les considérations financières priment la qualité de la prise en charge des malades. Les besoins spécifiques de chaque territoire ne sont pas pris en compte, si bien que, pour remédier au manque d'attractivité des carrières hospitalières, les hôpitaux doivent bien souvent faire appel à des intérimaires pour « boucher

Un plafonnement de ces rémunérations était prévu, mais il n'a toujours pas pu être mis en place, et pour cause : face à la pénurie de médecins, les hôpitaux, notamment les plus petits, ne peuvent pas se passer de l'intérim. la ministre : quand allons-nous changer de logique et faire passer l'intérêt des patients avant les intérêts financiers ? Quelle politique précise entendez-vous mettre en place pour restaurer durablement les carrières hospitalières et consolider notre système hospitalier ? La parole est à Mme la ministre

faciliter le développement de la télésanté. J'évoquerai enfin un autre axe d'action très important : nous sommes allés au-delà des frontières posées par les corporatismes pour pouvoir utiliser au maximum

il n'y a qu'à observer l'afflux massif de nos concitoyens pour se faire tester, l'augmentation démesurée des contaminations dans un temps record, ou la crainte pérenne pour beaucoup que cette période extraordinaire soit vouée à devenir ce qu'il y a de plus ordinaire. En coulisse, on voit des médecins, des urgentistes, des infirmiers, des ambulanciers, et j'en passe, épuisés et méprisés. La cinquième vague est là. Pourtant, l'hôpital va encore plus mal qu'au début de cette pandémie. Il meurt chaque jour un peu plus au gré de l'absence de décisions fortes et courageuses. À titre d'exemple, les professionnels médicaux et les soignants de l'hôpital d'Antibes ne cessent d'attirer mon attention sur la reconnaissance insuffisante du travail de nuit et la sous-valorisation de la permanence des soins, alors qu'ils sont au coeur de la bataille contre la covid-19, à l'exemple des services d'urgence, de réanimation ou encore de médecine. Certes, le Ségur de la santé a débouché sur un plan d'investissement dont nous ne pouvons que nous féliciter. Toutefois, l'hôpital français souffre d'un mal plus profond que la crise n'a fait que mettre en lumière. La multiplication des plans blancs, notamment dans mon département des Alpes-Maritimes, ne saurait masquer la multiplicité des défaillances dont l'hôpital est victime. Dès lors, plusieurs questions pourtant simples demeurent en suspens, madame la ministre. Qu'en est-il de la formation des infirmiers, alors qu'il est essentiel de « réarmer » les lits de réanimation- encore faut-il qu'il y en ait assez ! -occupés par nos concitoyens touchés gravement par le virus ? Comment expliquez-vous qu'en pleine pandémie ait été annoncé un retard dans la publication des décrets réformant les statuts et les conditions d'exercice des praticiens hospitaliers ?

question est en conséquence très simple : que comptez-vous faire pour éviter une saturation mortifère de nos hôpitaux à chaque pic épidémique ?

inconditionnel au directeur général du CHU de Guadeloupe et de ses collaborateurs qui ont été agressés hier soir au sein même de l'établissement public de santé. Je vous remercie de votre soutien, mes chers collègues.

Les nombreuses vagues de la crise sanitaire en outre-mer ont mis en évidence, davantage que dans l'Hexagone, les insuffisances structurelles de l'offre de soins dans ces territoires. En effet, les problématiques spécifiques de santé publique en outre-mer entraînent des surcoûts importants pour les établissements sanitaires et médico-sociaux.

quelles mesures entendez-vous prendre pour rétablir une équité salariale entre les différents personnels et garantir l'égalité d'accès à une offre de soins de qualité pour les usagers dans les outre-mer ? J'attends une réponse concrète.

à l'automne 2021 pour juger de l'opportunité et définir les conditions de mise en oeuvre d'une faculté de médecine de plein exercice aux Antilles. Aujourd'hui, les étudiants

L'ensemble des acteurs locaux ont été auditionnés par la mission, dont les conclusions seront remises au Gouvernement dans les prochaines semaines. Ainsi, nous pourrons déterminer rapidement le calendrier de mise en oeuvre de cette faculté de plein exercice aux Antilles. Madame la sénatrice, soyez assurée de notre détermination à faire aboutir ce projet,

que comptez-vous faire, notamment pour les Ehpad ?

pourtant tant attendus, sont à double tranchant. En effet, ils obligent contractuellement les établissements à réduire leurs dépenses sur une dizaine d'années, ce qui interdit tout nouvel emprunt.

Prenons l'exemple, dans mon département de la Savoie, du centre hospitalier de la vallée de la Maurienne. Le montant total des investissements nécessaires à la rénovation des services de médecine- stérilisation et blocs opératoires - s'y élève à 16,5 millions d'euros. Or une aide de 14,9 millions d'euros a bien été attribuée à l'hôpital dans le cadre du Ségur-

Cette aide est fournie dans le cadre d'une contractualisation avec l'ARS, définie par l'article 50 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et les décrets pris pour son application. Il y est précisé que chaque établissement bénéficiaire se verra fixer, au cas par cas, une trajectoire de désendettement, afin que l'objectif de restauration durable de sa santé financière soit respecté. Ces mesures sont prises pour que, à l'issue du Ségur, les établissements ne soient plus asphyxiés par leur dette, à la suite de nouveaux investissements insoutenables. En revanche, tous les endettements supplémentaires nécessaires à la réalisation réalisation des projets en cours d'instruction au moment de la contractualisation seront possibles. Je tenais à vous rassurer sur ce point : l'objectif est bien de poursuivre la transformation de l'offre de soins. Nous voulons simplement que cela ne se traduise pas par une course à l'endettement, qui menacerait à long terme la réalisation des projets des établissements. Dans le cas particulier que vous évoquez, et sans connaître les détails du dossier, je peux vous dire que tout endettement supplémentaire nécessaire à la réalisation du projet de rénovation soutenu par le Ségur sera pris en compte par l'ARS.

Comme l'écrit Edgar Morin, « à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel ». Le secteur médical, social et médico-social manifeste pour crier son désarroi devant des conditions de vie et de travail dégradées, mal reconnues ou indignes. Ils nous le à quoi bon continuer, alors qu'on est empêché de faire correctement notre travail ?». Le travail dans ces secteurs était difficile, il tend à devenir absurde au sens camusien du terme. Madame la ministre, le manque d'attractivité et la crise des vocations dans ce secteur se double aujourd'hui d'une fuite des personnels. Ces derniers démissionnent, sont en arrêt maladie, en invalidité, ou sont licenciés. Les jeunes quittent les métiers du secteur en moyenne au bout d'un an, voire au cours de leur formation. Des services entiers ferment, faute de personnel pour les faire tourner. Pendant ce temps, les besoins en termes de prise en charge des patients

L'ensemble des professions médicales et médico-sociales sont concernées, et ce problème ne fait qu'empirer malgré les nombreuses alertes. Aujourd'hui, le taux de vacance des postes dans mon département varie entre 15 %

de vie chère pourrait être versée aux soignants. En effet, le pouvoir d'achat en Haute-Savoie est faible pour les personnes qui travaillent en France, du fait de la proximité de la Suisse. Les revalorisations du Ségur de la santé n'ont pas permis et ne permettront pas de pallier le manque d'effectifs, les salaires suisses demeurant beaucoup plus avantageux. Une réflexion doit donc être menée conjointement avec la Suisse, afin de déterminer les actions pouvant être mises en place pour former plus de personnel et répondre aux besoins de nos pays. Il est également possible d'envisager une baisse des charges sociales et salariales, ce qui permettrait d'augmenter mécaniquement les salaires,

Monsieur le sénateur, les pénuries de personnel médical et médico-social en Haute-Savoie sont significatives, et je peux vous assurer que le Gouvernement y est particulièrement sensible.

Ces soignants ne viennent pas du Genevois français, mais de la France entière. Cet appel d'air est certes provoqué par les écarts de rémunération entre la Suisse et la France, mais aussi par le même phénomène de désaffection des métiers du soin, qui frappe aussi

sur laquelle les administrations centrales du ministère des solidarités et de la santé sont mobilisées. Il s'agit d'identifier les propositions susceptibles d'être adressées à nos partenaires suisses dans les prochaines semaines.

Meunier. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, « ne pas soutenir le soin, c'est ruiner la solidarité qui fonde l'État de droit ». C'est par ces mots empruntés à la philosophe Cynthia Fleury que je souhaite conclure ce débat. Si le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a choisi de consacrer cet espace de contrôle aux oubliés du Ségur de la santé, c'est qu'il lui semblait lui semblait que l'urgence de la situation sanitaire ne pouvait pas laisser à l'arrière-plan la question des conditions de travail, de carrière et de rémunération dans l'ensemble du secteur élargi des soins. L'alerte ne date pas d'hier, il est vrai. Les tensions dans les établissements sanitaires et médico-sociaux sont anciennes. Mais la crise sanitaire a mis en évidence la grande vulnérabilité de ces métiers et la grande fragilité de ces professionnels, qui risquent de raccrocher leur blouse à l'issue de la crise sanitaire, par désarroi ou par déconsidération. Récemment, les gestionnaires d'établissements parlaient même de « point de rupture

en dépit de la conférence des métiers de l'accompagnement social et du médico-social, initialement prévue pour le 15 janvier prochain et finalement reportée au premier trimestre 2022 en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, la patience des professionnels s'amenuise et les bénéficiaires en pâtissent.

les ambulanciers et les équipiers du SAMU dans les hôpitaux qui, auparavant alignés sur les aides-soignants, n'ont pas été reconnus comme étant au contact des patients. D'autres professionnels encore ont

On assiste alors à un nivellement par le bas, à la négation même des spécificités de ces métiers du soin, qui s'apprennent et dont les compétences et aptitudes sont sanctionnées par des diplômes d'État. Quel avenir réserve-t-on aux personnes faisant fonction d'aide-soignant ? Quelles sont les passerelles et les perspectives d'évolution ? Quel est le message envoyé aux personnels diplômés et aux rares jeunes qui se destinent à ce métier ? L'évolution des métiers du soin a fait l'objet de nombreux rapports qui devaient servir de fondement à une réforme ambitieuse du grand âge et de l'autonomie, mais je ne remuerai pas ici le couteau dans la plaie.

Permettre ainsi à des professionnels, à qui la société demande beaucoup, sur lesquels nous sommes reconnaissants de pouvoir nous appuyer lorsque nos proches ont besoin d'aide, ont besoin d'aide, de verbaliser leurs difficultés, leurs doutes, d'extérioriser les tensions accumulées, mais aussi de partager des moments de réussite et de progrès, est une manière incontournable de valoriser leur métier. Au-delà, je crois même que nous pourrions nous inspirer des pratiques dont Cynthia Fleury- encore elle -suggère l'application dans le secteur hospitalier. Elle propose des espaces de réflexion éthique, ouverts tant aux soignants qu'aux patients.

Vous le voyez, madame la ministre, mes chers collègues, la désaffection des métiers du « prendre soin » n'est pas inéluctable. Des pistes sont proposées. Elles méritent autant d'attention que ces professionnels en accordent chaque jour à nos proches. Voici